La séance est reprise. J'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Patrice Gélard, qui fut sénateur de la Seine-Maritime de 1995 à 2014. Un hommage lui sera rendu ultérieurement par M. le président du Sénat.

Le numérique apporte son lot d'opportunités nouvelles. Nous avons eu l'occasion de le vérifier au cours des derniers mois. La crise sanitaire nous a obligés à réinventer notre rapport à la culture et à l'éducation, à repenser nos moyens de communication et nos modes de travail. À bien des égards, c'est le numérique qui nous a permis de continuer à vivre en ces temps troublés. Cependant, il apporte également son lot de risques. Là encore, la période singulière que nous venons de vivre l'a rappelé le harcèlement en ligne n'a pas cessé, bien au contraire. J'en veux pour preuve la recrudescence des actes de pornodivulgation sur Snapchat- ce n'est qu'un exemple parmi d'autres des nombreuses menaces qui ont émergé avec le numérique. Face à ces menaces, nous avons une responsabilité : celle de faire respecter les règles par tous, de les adapter s'il le faut, de combler les vides juridiques afférents à ces nouveautés, avec pragmatisme, avec ambition, avec résolution, sans renoncer à nos principes et sans nous résigner. Ce n'est pas parce que les géants du numérique sont des « géants », en effet, qu'ils peuvent échapper à toute régulation. Non, internet n'est pas un espace de non-droit. Je veux vous le dire avec force : nous partageons le même état d'esprit. Nous ne pouvons pas nous contenter de ne rien faire alors que notre souveraineté est accaparée par des acteurs numériques étrangers. Il nous faut donc agir.

très bientôt l'occasion d'en parler avec les membres de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat. C'est ce même état d'esprit qui préside au texte que vous examinez aujourd'hui. Il étend à l'univers numérique une protection qui existe déjà pour les enfants du secteur du spectacle et les enfants mannequins.

de loi en est une preuve supplémentaire : la protection des enfants dans l'espace numérique est une priorité du Gouvernement, et nous sommes en train de renforcer Nous voulons notamment mieux protéger les mineurs contre la pornographie en ligne. La directive Services de médias audiovisuels y contribue. Elle impose aux plateformes de partage vidéo de mettre en place des mesures pour empêcher l'accès des mineurs aux contenus qui leur sont particulièrement préjudiciables, parmi lesquels figurent les contenus pornographiques. Elle sera rapidement La proposition de loi de la députée Bérangère Couillard, que vous avez adoptée à l'unanimité il y a deux semaines, va également dans ce sens. Elle a permis de préciser, dans le code pénal, que le simple fait de déclarer son âge en ligne ne constitue pas une protection suffisante contre l'accès des mineurs

les fournisseurs d'accès bloqueront la diffusion des sites concernés en France. C'est le moyen le plus efficace de protéger les mineurs. Un comité de suivi a en outre été mis en place pour encourager le recours au contrôle parental sur les terminaux, avec une obligation de résultat dans les six mois.

Je salue, en l'espèce, l'engagement de Roch-Olivier Maistre et de Sébastien Soriano, présidents respectivement du CSA et de l'Arcep, pour mener à bien cette coopération

Cette ambition, nous devons par conséquent la promouvoir au niveau européen, parce que l'Europe est notre meilleure protection- j'ai eu l'occasion de le dire à de multiples reprises à cette tribune. Face aux géants du numérique, elle est même notre seule protection efficace et crédible. Devant eux, nous ne ferons le poids que si nous faisons front commun. C'est le cas pour la question de la protection de l'enfance, comme c'était le cas pour la question du droit voisin, et comme cela sera évidemment le cas pour d'autres sujets à l'avenir. Justement, la Commission européenne prépare en ce moment même sa stratégie numérique. Elle vient de lancer une consultation publique sur la future législation relative aux services numériques, le, qui doit permettre de renforcer le marché commun et de clarifier les responsabilités en matière de services numériques. nous, une véritable occasion de promouvoir la vision française en la matière, par des initiatives ambitieuses concernant la régulation des contenus et la responsabilité des plateformes numériques. Je suis pleinement mobilisé, avec mon collègue Cédric O, secrétaire d'État chargé du numérique,

Cet engagement ne sera pas vain : il nous sera éminemment utile pour bâtir la régulation européenne de demain. Cette régulation devra être à la fois souple et exigeante. Souple, d'abord : le monde numérique change rapidement, et la régulation doit pouvoir changer tout aussi rapidement il faut donc fixer des objectifs, mais laisser les acteurs choisir les solutions les plus adaptées. Exigeante, ensuite ; cette exigence, nous l'atteindrons en dotant le régulateur de moyens pour contrôler les efforts et les résultats des plateformes, ainsi que pour sanctionner les manquements à leurs obligations.

sur YouTube principalement, mais aussi sur TikTok, Twitch ou, hier, Vine. Les plateformes de partage de vidéos sont, le plus souvent, une chance. Ce sont des espaces de liberté. Il s'y déploie une extraordinaire créativité. Des talents formidables s'y expriment, s'y révèlent, se trouvent un public, sans intermédiaires talents pour raconter des histoires, talents artistiques, musicaux, comiques ... Ces plateformes sont aussi une source de revenus pour les créateurs. Avec la monétisation des contenus, certains en ont même fait leur activité professionnelle- ils sont parfois qualifiés d'« influenceurs ». Néanmoins, aujourd'hui, de plus en plus de vidéos, de plus en plus de chaînes sont consacrées à l'exposition d'enfants.

cas échéant, imposent un rythme de tournage ou certains types de contenus ou de produits commerciaux. Ce sont les parents qui,, récupèrent la rémunération. Le risque pour les enfants est évident. Avec cette loi voulue par Bruno Studer, le président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, et par les députés, il s'agit de mieux protéger ces enfants « influenceurs ». Pour Pour protéger, il faut encadrer. Cela implique de faire entrer cette activité dans le droit commun du code du travail, pour le cas où l'activité des mineurs est assimilable au travail salarié. C'est déjà le cas- je le disais -pour les enfants qui jouent dans une pièce de théâtre, dans un film, ou qui font du cirque. Je salue d'ailleurs l'engagement de ma collègue Muriel Pénicaud en ce sens. Cela implique également de créer un régime de déclaration administrative, pour le cas où il ne s'agit pas de salariat, mais où le nombre et la durée des contenus ou le montant des revenus liés à la diffusion des vidéos justifient une vigilance particulière et une pédagogie auprès des parents. Pour protéger, il faut s'unir, associer les plateformes numériques à ce combat, les responsabiliser en matière d'information des parents sur la réglementation et de lutte contre les situations d'abus. Enfin, pour protéger, il faut garantir le droit à l'oubli. C'est ce que proposent les auteurs de cette proposition de loi pour les mineurs figurant sur des vidéos mises en ligne sur les plateformes numériques. Il importe tout particulièrement que le mineur n'ait pas besoin de demander l'autorisation de ses parents pour faire valoir ce droit. droit. Je tiens à remercier tous ceux qui ont travaillé à ce texte. Je remercie en particulier le président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, Bruno Studer, d'avoir déposé cette proposition de loi,

Tel est le sens des amendements que je souhaite vous soumettre au nom du Gouvernement ; l'un est rédactionnel, l'autre vise à préciser les règles applicables aux annonceurs afin de renforcer la réalité juridique du régime des sanctions, au regard notamment du principe de légalité des délits et des peines.

Il nous faudra aussi mobiliser les services de l'État pour détecter les situations particulièrement problématiques et garantir sans relâche la protection de l'enfance. Sur ce sujet, je peux vous assurer de la mobilisation pleine et entière du Gouvernement. La parole

la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui se situe à la convergence de deux préoccupations essentielles. La première d'entre elles est la protection des mineurs. Le travail des enfants est interdit dans notre pays depuis la loi de 1874. Pensons bien sûr aux de Victor Hugo ou à l'oeuvre de Charles Dickens, qui ont contribué, au XIX siècle, à l'éveil des consciences sur ce sujet. Les rares dérogations à ce principe, qui concernent les enfants du spectacle et du mannequinat, sont soigneusement encadrées par la loi. loi. Il faut bien le dire, l'enfance n'est pas le temps du travail et des préoccupations professionnelles. Si l'on peut concevoir une activité limitée, il nous appartient de préserver ce temps de l'insouciance. ce temps de l'insouciance. Or, si la révolution numérique a ouvert de nouveaux espaces de liberté et de créativité, ce dont il faut se réjouir, elle a également permis le développement de nouvelles formes d'exploitation, d'autant plus insidieuses qu'elles ont l'air parfaitement innocentes et ludiques. Il ne s'agit plus de travail « à la mine », certes, mais, depuis plusieurs années, les chaînes mettant en scène des enfants filmés par leurs parents se multiplient sur les plateformes de partage de vidéos en ligne. elles bénéficient, en France et dans le monde, d'une audience très importante, qui peut atteindre plusieurs millions d'abonnés et des dizaines de millions de vues.

Comment croire, dès lors, à la fiction soigneusement entretenue de vidéos tournées et produites de manière « naturelle », sans pressions ni contrainte ? Quand des sommes aussi considérables que celles qui ont été évoquées durant les auditions- parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois ! -sont en jeu, comment penser une seule seconde que l'équilibre de ces enfants est préservé ?

Le grand mérite de la proposition de loi de Bruno Studer, président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, qui a été adoptée à l'unanimité par les députés, est de commencer à constituer un cadre juridique qui réponde à ces nouveaux défis.

Protéger : tel est, en un mot, l'objet de la présente proposition de loi, qui s'inscrit dans un mouvement amorcé depuis déjà plusieurs années, consistant à réguler internet pour éviter que celui-ci ne soit un espace de non-droits, « sans foi ni loi ». C'est là un exercice délicat pour le législateur, qui doit mettre en balance la sauvegarde des libertés publiques, au premier rang desquelles figure la liberté de communication, et la protection du « vivre ensemble » et des plus vulnérables. La récente décision du Conseil constitutionnel sur la proposition de loi Avia visant à lutter contre la haine en ligne nous a montré, si besoin était, qu'il fallait suivre un chemin de crête particulièrement étroit et que l'on a toujours intérêt à écouter très attentivement, en la matière comme en bien d'autres, les justes préconisations de Philippe Bas, éminent président de la commission des lois du Sénat. Je souhaite attirer votre attention sur trois points qui font, selon moi, la pertinence de ce texte. En premier lieu, cette proposition de loi prend en compte la nature profondément mouvante de l'espace numérique

des vidéos « amateurs » et de celles, enfin, qui s'inscrivent aujourd'hui dans une « zone grise », jouant sur la porosité des frontières entre travail et loisir. Plusieurs régimes juridiques sont définis pour s'adapter au mieux à la diversité des situations rencontrées. Ce souci du réel se retrouve aussi dans la disposition qui élargit le fameux « droit à l'oubli ». Les mineurs pourront désormais exercer ce droit sans le consentement de leurs représentants légaux, lesquels peuvent avoir un intérêt au maintien de certains contenus en ligne. En deuxième lieu, cette proposition de loi a le mérite de placer chaque acteur face à ses responsabilités, ce qui n'est pas superflu. Les parents, tout d'abord, sont les premiers responsables non seulement de ces vidéos, mais surtout de la sauvegarde du bien-être de leur enfant. Hélas, ils sont encore trop nombreux à ne pas mesurer les risques d'une telle exposition de l'image de leur enfant sur internet, d'où la nécessité et l'urgence de mieux éduquer l'ensemble de la société aux enjeux du numérique- sujet cher à notre présidente Catherine Morin-Desailly. Je salue d'ailleurs l'excellente initiative de notre collègue Sylvie Robert, qui propose, par un judicieux amendement, d'élargir les obligations de sensibilisation des plateformes en direction des mineurs eux-mêmes.

Celles-ci auront pour obligation d'adopter, sous le contrôle du CSA et de Roch-Olivier Maistre, des chartes destinées par exemple à favoriser la mise en place de procédures de signalement par les utilisateurs des contenus problématiques portant atteinte à la dignité ou à l'intégrité d'un mineur. Soulignons enfin que, si ce texte n'a vocation à s'appliquer qu'à une minorité d'enfants et de parents, sa portée symbolique est considérable.

Lors de ses travaux, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat a veillé en particulier à la qualité rédactionnelle du texte et s'est attachée à préciser certains points dans le sens d'une meilleure garantie des droits des mineurs. Dans un souci de transparence et de pédagogie, il nous a également semblé essentiel d'assurer aux parents une meilleure information sur le contenu de leurs obligations financières- je remercie une nouvelle fois notre collègue Laurent Lafon pour ses amendements en ce sens.

J'entends les interrogations qui subsistent quant à l'effectivité du texte. Il appartiendra certainement à la jurisprudence d'affiner, au fur et à mesure, les distinctions entre ces nouveaux régimes juridiques. cette proposition de loi est- j'en suis intimement persuadé -la solution la plus convaincante dont nous disposons à ce stade.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,

Je citerai l'examen de la proposition de loi relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique et le débat sur la proposition de loi visant à lutter contre l'exposition précoce des enfants aux écrans, déposée par la présidente de la commission de la culture du Sénat. Aujourd'hui, nous sommes conduits à discuter de l'exploitation commerciale des vidéos mettant en scène des mineurs de moins de 16 ans mises en ligne sur des plateformes de partage telles que YouTube. Dans leur finalité, les différents textes précités se rejoignent : ils ont pour objet de protéger les enfants en tenant compte de l'évolution des usages, et singulièrement des usages numériques. Après l'euphorie des premières années internet, nous avons collectivement pris conscience que l'entrée dans la « troisième révolution industrielle » s'accompagnait d'enjeux auxquels il s'avérait absolument impératif d'apporter des réponses : protection des données,

en effet des questions aiguës concernant les droits des mineurs. Notre ordre juridique interne, reposant sur le postulat selon lequel ses représentants légaux agissent au nom du mineur, n'est pas suffisamment opérant ni approprié pour appréhender l'ensemble des usages numériques et protéger ainsi efficacement les mineurs.

peut s'opposer à ce que les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale aient accès aux données le concernant recueillies au cours [de projets de recherche] ». L'article 5 de la présente proposition de loi est une autre illustration probante d'une telle évolution, puisqu'il confère aux mineurs un droit à l'oubli sans que le consentement des titulaires de l'autorité parentale soit requis.

proposition de loi comble un vide juridique afférent à une pratique de plus en plus courante : la réalisation et la publication de contenus mettant en scène des enfants sur des plateformes en ligne.

effet indispensable de porter une vive attention aux risques, notamment psychologiques, inhérents aux conditions et à la fréquence de production de ces vidéos, mais aussi- vous l'avez dit, cher rapporteur -au respect de la dignité physique et morale de ces enfants, en veillant à ce que les contenus mis en ligne n'y portent aucunement atteinte. Cependant, étrangement, cette sensibilisation, essentielle, qui passe notamment par la responsabilisation des plateformes, lesquelles devront édicter des chartes, ne s'adresse pas aux principaux acteurs concernés, c'est-à-dire aux mineurs eux-mêmes. Pourtant, il s'avère fondamental de faire preuve de pédagogie à leur égard, dans un souci d'éducation, de responsabilisation et de protection. C'est pourquoi nous proposons d'informer et d'alerter ces mineurs sur les conséquences de la diffusion de leur image, tant sur leur vie privée

qui réalisent et diffusent par eux-mêmes des vidéos- ils sont nombreux dans ce cas -sans avoir nécessairement conscience des risques qui en découlent. Cette logique alliant pédagogie et responsabilisation est pertinente

Nous le voyons, mes chers collègues : sur tous ces sujets, notre droit est en construction. Souhaitons qu'il soit respecté par tous, mais n'oublions pas que, face à la « perfusion numérique » et

depuis la diffusion large de l'internet, à compter du début des années 2000, l'usage qui en est fait soulève fréquemment de nouvelles problématiques. Cet espace de création et d'expression, qui s'affranchit volontiers des frontières, connaît naturellement aussi ses dérives et ses excès.

comme le rappelle souvent Mme la présidente Catherine Morin-Desailly au sein de notre commission. Le législateur français a pu en faire aisément le constat lorsqu'il a souhaité s'emparer de problématiques relatives à l'encadrement de l'expression au sein de ce nouvel espace. La majorité présidentielle a ainsi, à plusieurs reprises depuis le début de la législature, déjà entrepris d'apporter des réponses, qu'il s'agisse de lutter contre la manipulation de l'information ou contre la diffusion de contenus haineux. Dans le premier cas de figure, sur la majorité des travées de cet hémicycle, nous avons estimé que l'objectif visé n'était pas correctement ciblé par les nouvelles dispositions introduites par les députés de la majorité et que ces dernières pouvaient même,, s'avérer pernicieuses. Dans le second cas de figure, c'est le Conseil constitutionnel lui-même qui a censuré le principal apport du texte, pointant que l'obligation faite aux réseaux sociaux de supprimer dans les vingt-quatre heures, sous peine de lourdes amendes, les contenus « haineux » qui leur sont signalés risquait de porter une atteinte à l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée ». C'est cette fois sur l'initiative de M. le président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, soutenu dans sa démarche par le groupe LaREM, que nous sommes amenés à réfléchir à l'encadrement de l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne. Ces dernières, telles que YouTube, hébergent des chaînes sur lesquelles des mineurs de moins de 16 ans sont mis en scène, la plupart du temps par des membres de leur famille, l'ambition créatrice des

L'intention du législateur, au travers de ce texte, est, d'une part, de faire bénéficier les mineurs filmés des garanties prévues pour les enfants du spectacle en matière de temps de travail et de rémunération, et, d'autre part, de prévenir les conséquences psychologiques de long terme susceptibles d'affecter ces enfants. Le groupe RDSE partage pleinement la préoccupation de l'auteur de la proposition de loi. Il nous faut globalement mieux appréhender l'éducation au numérique des jeunes générations, mais également celle des moins jeunes. La prévention peut et doit, par le biais notamment, dans les années à venir, de l'action d'enseignants pour lesquels ce type d'outils sera sans doute plus familier, permettre une utilisation plus raisonnée et modérée de l'internet chez beaucoup d'entre nous, notamment les plus jeunes. Ces derniers, tout comme leurs parents, doivent pouvoir mieux appréhender les conséquences, tout particulièrement psychologiques, qui peuvent être liées à une surexposition de leur image sur la « toile Cette mobilisation pour donner à chacun les meilleures clés de compréhension d'un outil numérique capable de broyer des individus nous paraît toujours aussi indispensable. Nous saluons donc l'initiative du président Studer, qui propose d'instaurer un cadre légal équilibré et pionnier en la matière, en opérant notamment un distinguo entre vidéos professionnelles, vidéos semi-professionnelles et vidéos amateurs, et en soumettant chacune de ces catégories à un cadre juridique spécifique. La responsabilisation voulue par le législateur porte en outre sur les parents, mais également sur les entreprises susceptibles de conclure des contrats de placement de produits, ainsi que sur les plateformes accueillant ces vidéos. Nous saluons aussi le travail approfondi de notre rapporteur qui, par des précisions opportunes et un renforcement des contraintes appelées à peser sur les plateformes, est venu affiner le caractère opérationnel de cette proposition de loi. égard aux remarques formulées au début de mon intervention sur l'impérieuse nécessité de trouver une réponse internationalement concertée, au moins à l'échelon européen, qui soit la plus à même d'imposer aux géants de l'internet des garde-fous, nous sommes tentés d'émettre des réserves sur-la portée véritable de ce texte. Toutefois, cette proposition de loi nous apparaît pertinente et équilibrée sur le plan du droit.

Nous soutiendrons donc cette initiative qui permet de poser clairement le débat, un débat essentiel puisqu'il a trait à la protection de l'enfance en matière numérique. Le groupe RDSE votera la présente proposition de loi.

très chaleureusement notre collègue et ami Jean-Raymond Hugonet pour le travail de grande qualité qu'il a réalisé dans des délais, disons-le, particulièrement courts. Le fait qu'il ait été désigné rapporteur et, surtout, son approche résolument constructive de l'examen du texte en commission témoignent du caractère éminemment transpartisan de cette proposition de loi. Je trouve personnellement essentiel que nos deux chambres, quelle que soit leur coloration politique respective, soient capables d'oeuvrer en pleine syntonie lorsqu'il y va de la protection de nos enfants, de leur épanouissement et de leur santé mentale. La soumission à une mode d'un jour qui perdure dans le temps pour devenir le symbole d'une génération ne doit pas nous faire oublier « la cause des enfants », pour reprendre le titre d'un des plus fameux ouvrages de Françoise Dolto. Il y a maintenant quinze ans apparaissaient pour la première fois, sur les plateformes de partage de vidéos nouvellement créées, des vidéos mettant en scène des enfants dans leur vie quotidienne. Il y a quelques années, partout dans le monde, de jeunes enfants, à l'instar du désormais célèbre Ryan Kaji, commençaient à être filmés presque quotidiennement par leurs parents, les vidéos ainsi réalisées totalisant des millions, parfois même des milliards, de visionnages. L'année dernière, le « jeter de fromage » au visage de bébés, provoquant souvent, hélas ! l'hilarité des parents qui les filment, est devenu un phénomène viral sur ces mêmes plateformes et sur les réseaux sociaux. Il faut d'ailleurs rappeler que ce type de vidéos prétendument novateur n'est en réalité qu'une reprise au goût du jour, pour ne pas dire au mauvais goût du jour,

Ce vide juridique qu'il faut combler et ces dérives qu'il faut empêcher nous renvoient, nous, parlementaires, à notre responsabilité de législateur. Le législateur est pleinement dans son rôle pleinement dans son rôle lorsqu'il met en lumière des situations de travail qui demeurent inconnues de nombre de nos concitoyens. Il est dans son rôle quand il s'agit d'étendre le régime protecteur des enfants du spectacle et de la mode aux enfants dits « youtubeurs » et lorsqu'il place les plateformes face à leurs responsabilités en les contraignant au retrait des contenus lorsque les diffuseurs de ces derniers font fi de l'obligation d'autorisation préalable. Il est également dans son rôle, chers collègues, quand il instaure un droit à l'oubli que les mineurs peuvent solliciter pour obtenir le retrait des vidéos où ils apparaissent.

En somme, vous l'aurez compris, le législateur est dans son rôle quand il protège ! J'aimerais d'ailleurs, à ce titre, rappeler combien ce texte est consubstantiel de l'esprit qui anime notre République, la République des droits de l'homme, la République qui protège les plus fragiles, la République qui montre le chemin à suivre aux autres pays quand il s'agit de garantir les droits de chacun, particulièrement des plus vulnérables. La France est en effet le premier pays au monde à s'emparer de ce sujet. La France

enfants. J'entends dire, ici et là, que cette proposition de loi ne sanctionne pas assez, qu'elle ne résout pas tous les problèmes. À cela, je réponds que l'avènement du monde numérique et des plateformes de partage de vidéos a engendré une myriade de problèmes que nous ne réglerons pas d'un seul coup, que

de ce texte innovant qui constituera, espérons-le, la première pierre d'un édifice plus vaste et plus protecteur encore, qu'il nous faudra bâtir ensemble.

Ce vide juridique les expose à des abus, y compris de la part de leurs parents, qui ne maîtrisent pas toujours les dérives liées à la diffusion de ces vidéos. Plusieurs risques doivent être écartés. Parmi les plus graves figurent les commentaires haineux, l'agressivité et le cyberharcèlement, qui peuvent avoir des conséquences dramatiques sur leur santé mentale. Des adolescents sont poussés au suicide par la violence des réseaux sociaux. Nous avons le devoir de prévenir ces tragédies. Un autre risque doit nous inquiéter, celui du décrochage éducatif. Tous les parents sont aujourd'hui confrontés aux excès dans l'usage du numérique par les adolescents. Le contrôle parental est devenu un combat quotidien, dans lequel les adultes sont de plus en plus démunis, faute de moyens. Là encore, il faut poser des limites, pour éviter que ces enfants ne s'éloignent de la vie scolaire en consacrant un temps excessif aux plateformes en ligne. Enfin, le traitement des questions relatives aux conditions de travail et aux revenus engendrés par ces activités constitue un pilier essentiel de la future loi. Ce pilier législatif a été largement enrichi par la commission de la culture du Sénat, qui a précisé les responsabilités légales des parents, à la fois « employeurs » et propriétaires des chaînes YouTube de leurs enfants.

cette proposition de loi vise à combler le vide juridique dans lequel se trouve aujourd'hui l'exploitation commerciale des enfants sur les plateformes numériques. C'est un premier pas que nous saluons,

qui ont pourtant une audience, des salariés et des utilisateurs, parfois même professionnels, dans notre pays, sont nombreuses. Cela doit nous amener à redéfinir aussi la fiscalité à laquelle sont soumis les Gafam et YouTube. Chacun sait en effet que le montant des taxes qu'ils acquittent est bien en deçà de ce que l'on pourrait imaginer. Ces plateformes numériques doivent contribuer au financement de la création, puisqu'elles en tirent des ressources colossales. L'enjeu central de cette proposition de loi est de faire respecter les droits de l'enfant. est très complexe, nous en avons tous conscience. Cela implique de les protéger des rythmes effrénés de tournage qui leur sont parfois imposés et de contrôler si les contenus dans lesquels ils figurent sont compatibles avec leur âge. Cela nécessite aussi de réexaminer la nature de ces nouvelles pratiques et leur compatibilité, par exemple, avec l'obligation scolaire. Être filmé déballant des cadeaux d'anniversaire ou visitant un parc d'attractions pourrait devenir du travail déguisé. Cette question du travail caché derrière des activités ludiques est primordiale,

les commentaires et les réactions de « spectateurs ». Se pose enfin la question de l'« après », quand l'enfant-star devient adolescent ou adulte. L'émergence des plateformes marque l'avènement d'une société où le « succès » arrive aussi vite qu'il repart. Chacun mesure les dommages que cela peut causer sur des esprits en construction. Nous devons continuer à nous interroger collectivement et à construire des réponses concrètes en termes de protection des enfants et des jeunes. C'est un sujet de réflexion dont aurait pu s'emparer la délégation aux droits des enfants que notre groupe avait proposé de créer au Sénat.

Face à ce constat, un acteur doit se réaffirmer avec force : le service public. Qu'il offre une alternative éducative, ludique et culturelle, et nous ferons vivre l'exception culturelle française

la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui s'inscrit dans la lignée des récentes dispositions adoptées par le Parlement visant à adapter notre législation aux évolutions rapides de notre société.

au monde numérique. Ce processus de mise à jour de notre corpus juridique demande une attention soutenue pour ne laisser aucun domaine sans protection. La proposition de loi « visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne » offre des réponses

à un âge où les principaux intéressés ne sont pas en mesure d'apporter un consentement éclairé à la diffusion de leurs faits et gestes auprès de millions d'abonnés dans le monde entier, qui plus est lorsqu'il s'agit de faire la promotion d'un produit ou d'une marque. Qu'il s'agisse de vidéos monétisées ou visant au placement de produits, certaines situations seraient qualifiables de travail illicite d'enfants, d'autres pourraient donner lieu à des poursuites pour maltraitance. Par ailleurs, nous connaissons encore mal l'impact psychologique d'une exposition aussi précoce, régulière et massive de la vie privée d'un enfant aux regards de tous. Nous sommes d'ores et déjà conscients du risque de cyberharcèlement auquel les enfants filmés sont exposés. L'autre versant de la question qu'il nous faut considérer, c'est l'impact de ces nouveaux modèles auxquels s'identifient des millions d'enfants. Leurs héros ne sont plus des personnages de la littérature pour

La culture du livre se fonde sur une recherche de sens au moyen de la narration. La culture des écrans, elle, repose sur la délivrance immédiate d'une information disponible de façon illimitée. Le passage brutal de l'une à l'autre inquiète un certain nombre de chercheurs, qui craignent l'émergence d'une génération sans repères et sans discernement. Un certain nombre de dérives et d'incertitudes existent. Il est grand temps de dissiper le flou législatif qui entoure la diffusion de vidéos de mineurs sur des chaînes familiales.

Tout d'abord, l'article 1 vise à étendre le cadre juridique applicable aux enfants du spectacle aux enfants dont l'image est exploitée commercialement sur les plateformes. Ce cadre prévoit un encadrement des durées et conditions de travail, une demande préalable d'autorisation, ainsi que l'ouverture d'un compte à la Caisse des dépôts et consignations. à mettre en place un dispositif intermédiaire entre le statut amateur et le statut professionnel de parent producteur. Il s'agit d'un cadre semi-professionnel, prévoyant une limitation de la durée des activités à laquelle le mineur participe, ainsi qu'un partage des revenus générés. Ce statut s'appliquera lorsque l'activité en question dépassera un certain seuil en termes de durée ou de rémunération. Autre avancée importante de cette proposition de loi, l'article 5 vise à étendre l'exercice du droit à l'oubli aux mineurs.

Je souhaite remercier le rapporteur, Jean-Raymond Hugonet, de son travail, en particulier sur l'article 2, qui tend à conférer au juge judiciaire la possibilité d'ordonner le déréférencement des vidéos illégales sur signalement de l'administration. cette proposition de loi est une occasion importante de renforcer notre législation en matière de protection de l'enfance. Notre groupe y est favorable.

comparaison,, le numéro un au, comptabilise 20 millions d'entrées. Cela permet de mettre en perspective la publicité et les revenus que peuvent générer de telles activités.

je veux parler du cinéma, du théâtre, du cirque, de la danse, de l'art vivant en général, mais aussi du mannequinat -, doivent l'être également, et même surtout, quand

J'ai à l'esprit l'exemple d'une jeune fille qui s'enregistrait régulièrement sur TikTok, plateforme sur laquelle des jeunes reproduisent des chorégraphies. Elle a été victime de harcèlement et a dû arrêter ses vidéos.

Je m'éloigne du sujet de cette proposition de loi, me direz-vous ? Et pourtant ... Le seul fait d'évoquer TikTok nous amène au coeur du sujet

ne suffisait pas. Je considère qu'il faut donner ce pouvoir au CSA, mais je redoute que l'on ne découvre rapidement qu'un juge français n'a pas grand pouvoir sur une multinationale dont le siège est implanté bien Une nouvelle fois, ce sujet nous renvoie à la nécessité de traiter la question de la souveraineté numérique au niveau européen, comme vous l'avez rappelé, monsieur le ministre. Cette réflexion européenne a d'ailleurs débuté, elle a même déjà donné de premiers résultats, mais la route est encore longue, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas la poursuivre. À ce titre, nous vous remercions de votre engagement, monsieur le ministre. Pour autant, ce texte est utile ; il comporte de très bonnes mesures. Je pense à la création de statuts spécifiques pour encadrer l'exploitation de l'image des mineurs, à savoir un statut professionnel et un statut semi-professionnel correspondant assez bien aux pratiques des créateurs de contenus sur les plateformes numériques.

la sécurisation des revenus et à la garantie que les enfants bénéficieront, à leur majorité, du fruit de leur travail. Je salue, au passage, l'amendement de mon collègue Laurent Lafon visant à améliorer l'information des parents à ce sujet.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, parfois la loi anticipe, parfois elle s'adapte. Dans le domaine du numérique, pour de multiples raisons notamment liées à la protection de la liberté d'expression et à la mondialisation, force est de constater que la législation a un retard considérable sur l'innovation. YouTube a été créé en 2005, a atteint le milliard d'abonnés en 2010 et compte plus de 2 milliards d'utilisateurs en 2020. Chaque minute, plus de 300 heures de vidéos sont mises en ligne. Chaque mois, plus de 1 milliard d'utilisateurs uniques se connectent à YouTube et visionnent près de 6 milliards d'heures de vidéo. Parmi les chaînes YouTube ayant produit le plus de revenus en 2019, on compte celles de deux enfants de moins de 8 ans. À eux deux, ils auraient perçu près de 44 millions de dollars en un an. Que ce succès soit le fruit d'un accidentel, d'une opportunité exploitée ou d'un élaboré, la diffusion de vidéos constitue désormais une activité professionnelle à part entière pour ces deux enfants. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui constitue donc une avancée indispensable en la matière, en ce qu'elle vise à encadrer l'exploitation commerciale de l'image des mineurs. Je remercie mon collègue Jean-Raymond Hugonet pour son travail et son implication en tant que rapporteur, ainsi que l'ensemble de la commission, très mobilisée sur ces sujets. L'article 1 crée, pour les mineurs de moins de 16 ans, le cadre légal d'exercice de la profession d'« influenceur » sur l'ensemble des plateformes en ligne. Il s'agit d'une avancée considérable pour la reconnaissance de la professionnalisation de cette activité, mais aussi et surtout en matière de lutte contre le travail dissimulé des mineurs. Les dispositions relatives à l'information des parents sur les droits de l'enfant, les modalités de réalisation des vidéos et les conséquences de l'exposition de son image sont également essentielles et leur effectivité sera, je l'espère, appuyée par la nouvelle mission attribuée au CSA par l'article 4. L'article 3 constitue également une avancée importante, puisqu'il pose les bases législatives permettant de dissocier l'usage récréatif de l'usage professionnel des plateformes en ligne pour les mineurs de moins de 16 ans, tout en garantissant la protection de leurs revenus. L'article 5 vient compléter le droit à l'oubli en précisant son application stricte, sans condition de consentement des titulaires de l'autorité parentale, pour les mineurs. Par là même, il répond à une problématique de plus en plus récurrente dans le monde entier.

d'un cadre pénal fixant les sanctions d'un délit d'atteinte reposant sur la présomption de consentement me semble indispensable à l'avenir. Ce mécanisme imposerait de rendre les parents pénalement responsables de la protection de la vie privée de leurs enfants mineurs.

mais également en cas d'atteinte à la vie privée d'un autre mineur commise par leur enfant ? La réponse me semble comprise dans la question. Alors que la dictature de l'image devient omniprésente dans la vie des des enfants, et ce dès leur plus jeune âge, que nous assistons à une progression fulgurante de troubles mentaux et comportementaux liés à l'anxiété qui en découle- je pense au phénomène du cyberharcèlement

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis plusieurs années, les « chaînes » mettant en scène des enfants se multiplient sur les plateformes de partage de vidéos en ligne. Elles sont souvent réalisées et diffusées par des membres de la famille. Ces nouvelles pratiques rencontrent un succès croissant en France comme à l'étranger. De nombreuses questions se posent en termes d'éthique quant au contenu des vidéos, aux heures de tournage ou aux revenus produits. La proposition de loi de notre collègue député Bruno Studer, que je salue, vise à combler le vide juridique existant, en mettant en place un cadre légal protecteur, pour les enfants de moins de 16 ans acteurs de vidéos diffusées sur des plateformes en ligne, de l'exploitation de leur image sur internet. Je tiens à remercier et à féliciter notre collègue rapporteur Jean-Raymond Hugonet, dont le rapport pose bien les enjeux sur ce sujet essentiel. Cette proposition de loi offre des garanties en matière de durée du travail des enfants et de protection de leurs revenus ; c'est l'objet de l'article 1.

qui participent à des vidéos partagées sur des plateformes, mais qui ne relèvent pas des procédures d'autorisation ou d'agrément prévues par le code du travail. L'article 5 autorise les mineurs à exercer eux-mêmes le droit à l'effacement des données institué par le règlement général par un service de plateforme de partage de vidéos, y compris dans le cas où leurs représentants légaux s'y opposeraient. C'est une avancée salutaire. Je concentrerai mon propos sur l'article 4, qui introduit l'obligation, pour les services de plateforme de partage de vidéos, d'adopter des chartes ayant notamment pour objet de favoriser le signalement, par leurs utilisateurs, de contenus qui porteraient atteinte à la dignité ou à l'intégrité morale ou physique des enfants et d'améliorer, en lien avec des associations de protection de l'enfance, la détection de situations qui porteraient atteinte à la dignité ou à l'intégrité morale ou physique des mineurs. En 2019, dans le cadre de la mission commune d'information sur les politiques publiques de prévention, de détection, d'organisation des signalements et de répression des infractions sexuelles susceptibles d'être commises par des personnes en contact avec des mineurs

comme la découverte de sites hébergeant des millions de photos d'enfants, récupérées sur les réseaux sociaux puis classées dans des catégories ne laissant guère de doutes sur le caractère pédophile de la plateforme et son activité criminelle.

Comme le précise Interpol, en matière de lutte contre la pédocriminalité, le meilleur moyen de protéger nos enfants est d'entretenir un dialogue franc et ouvert avec eux sur l'utilisation des médias sociaux, des applications, des jeux vidéo et d'internet. Il faut les sensibiliser aux dangers d'internet dès que possible, idéalement dès qu'ils commencent à le protection des enfants est de la responsabilité des plateformes, des entreprises de placement de produits, mais aussi des parents. Ce texte a fait l'objet d'évolutions lors de son examen à l'Assemblée nationale et a été largement amélioré par notre commission de

en renforçant la sécurité juridique des parties concernées. Il s'agit de s'aligner sur le régime de droit commun prévu par le code du travail. L'amendement prévoit ainsi que les annonceurs devront vérifier auprès des parents si l'obligation de consignation des revenus s'applique.

La séance est reprise. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun. demande du groupe La République En Marche, de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l'arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent

en deuxième lecture. Cette proposition de loi part d'un constat : en France, 3 % ou 4 % seulement des victimes d'arrêt cardiaque survivent, alors que ce taux est bien plus fort- il peut atteindre 40 % -dans certains pays anglo-saxons ou scandinaves. Comment expliquer cette différence ? Plusieurs facteurs peuvent entrer en jeu, mais l'un d'entre eux est incontestablement la formation insuffisante des Français aux gestes qui sauvent.

Nous sommes pleinement conscients de cet enjeu ; c'est la raison pour laquelle le Président de la République s'est engagé à ce que 80 % de la population soit formée aux premiers secours dans un délai de dix ans. C'est un délai raisonnable, mais exigeant. Il appelle tous les acteurs- administrations, entreprises, associations -à travailler ensemble et il invite à former à tout âge. Nous nous y attelons depuis le début du mandat, et nous n'avons pas l'intention d'arrêter. Notre objectif est d'améliorer le taux de survie en cas d'arrêt cardiaque en le faisant passer à 10 %, ce qui permettrait de sauver 3 000 vies par an. Aussi la multiplication prévisible des interventions de citoyens pour prêter assistance à des victimes méritait-elle une attention particulière et devait-elle être prise en compte dans la loi.

ce statut est également un signal, une garantie, une protection supplémentaire pour toutes celles et tous ceux qui pratiqueraient les premiers secours sur une victime, en ce que les citoyens sauveteurs seront exonérés de toute responsabilité civile, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle. Ce texte comporte également d'autres avancées. Par ses dispositions relatives à la formation à l'école, il s'inscrit dans la droite ligne de l'action engagée par le Gouvernement. Cette année, 80 % des élèves de troisième devaient recevoir une formation aux premiers secours, et 100 % des élèves devraient être formés dès l'année dès l'année prochaine. J'ajoute que le service national universel (SNU) sera l'occasion de renforcer la formation de notre jeunesse aux gestes qui sauvent. L'article 4 du texte, quant à lui, répond à un enjeu de poids en permettant de garantir la formation et la sensibilisation à tous les âges, y compris en milieu professionnel. La proposition de loi instaure également une journée nationale de lutte contre l'arrêt cardiaque, qui permettra de renforcer l'attention de chacun à cette question et d'inciter encore davantage de Français à se former. Enfin, le texte permet de renforcer les pouvoirs de contrôle du Parlement. C'est une bonne chose, et je suis satisfait que le Parlement puisse disposer des éléments utiles pour évaluer les résultats de notre action dans cette lutte si nécessaire contre les arrêts cardiaques. Mesdames, messieurs les sénateurs, ce texte fait, je crois, l'objet d'un large consensus, que nous devons saluer. Il permet des avancées, notamment une meilleure protection des Français qui interviendraient pour sauver des victimes. Il offre l'assurance d'une attention plus forte à la question des arrêts cardiaques et répond aux enjeux de la formation aux premiers secours en milieu scolaire ou en milieu professionnel.

monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui en deuxième lecture la proposition de loi relative au statut de citoyen sauveteur, sur laquelle nous nous étions déjà penchés au mois d'octobre dernier. Pour rappel, cette proposition de loi a été déposée sur l'initiative de notre collègue député Jean-Charles Colas-Roy, membre du groupe La République En Marche de l'Assemblée nationale, qui est également rapporteur de ce texte. Par le biais de diverses mesures, la proposition de loi vise à faire décroître le taux de mortalité très important des arrêts cardiaques en France. En première lecture, le Sénat avait naturellement souscrit à cet objectif, mais une analyse juridique scrupuleuse avait conduit la commission des lois à supprimer sept des douze articles que comportait le texte transmis. En effet, les dispositions que tendaient à introduire ces articles n'entraient pas dans le champ matériel que l'article 34 de notre Constitution confie à la loi. En outre, certains de ces articles étaient déjà satisfaits par les règlements en vigueur. Le superflu ayant été ôté, nous nous étions attelés à parfaire la rédaction et l'efficacité des dispositions restantes. Ainsi, nous avions récrit l'article 1, relatif au régime de responsabilité civile et pénale du sauveteur. Nous avions également précisé la rédaction de l'article 11, tendant à inscrire dans le code pénal des circonstances aggravantes pour le vol ou la détérioration de matériels de secours. Nous avions également profité du dispositif de l'article 7 pour autoriser certains personnels de santé, dont la liste sera fixée par décret, à accomplir les actes de sensibilisation au secourisme aux côtés des acteurs de la sécurité civile. C'est donc un véhicule bien plus léger, mais beaucoup plus efficace, que nous avions renvoyé à l'Assemblée nationale pour examen en deuxième lecture. Le texte qui nous parvient aujourd'hui atteste que notre démarche a été comprise par nos collègues députés, lesquels ont conservé la majeure partie des modifications que nous avions apportées.

positif et sans lien avec l'objet de la présente proposition de loi. La commission des lois maintient sa position à ce sujet, mais elle considère qu'il ne s'agit pas d'une malfaçon rédhibitoire, rédhibitoire, depuis que le rapporteur de l'Assemblée nationale a clarifié, dans son rapport, la manière dont le terme « citoyen » doit être entendu s'agissant de ce texte. La seconde modification réside dans la réintroduction du détail des diligences devant être mises en oeuvre par le citoyen sauveteur portant assistance à la victime d'un arrêt cardiaque. Nous avions supprimé cette mention, considérant que son exhaustivité pourrait décourager les sauveteurs à agir. Ici aussi, la commission des lois maintient sa position et regrette cette réintroduction, mais elle n'entend toutefois pas en faire un grief insurmontable. Les suppressions ou adoptions conformes de six articles dans la version du Sénat sont aussi à compter au nombre de nos satisfactions, mais tous les articles écartés par le Sénat en première lecture n'ont pas connu ce destin, heureux selon nous, puisque quatre d'entre eux ont été réintroduits par l'Assemblée nationale. Ainsi, les articles 2 et 4, relatifs respectivement à la sensibilisation des élèves au secourisme et au droit à la formation aux premiers secours pour tout salarié,

Il en va de même de l'article 6, tendant à créer une journée nationale de lutte contre l'arrêt cardiaque, réintroduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Je maintiens que la création d'une journée nationale n'est pas du domaine de la loi et que de nombreuses journées de ce type existent déjà. Enfin, l'Assemblée nationale a réintroduit l'article 12 , qui enjoint au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport annuel. Nul besoin de vous rappeler, chers collègues, la position du Sénat à ce sujet La commission des lois considère que ces réintroductions, si elles ne sont pas souhaitables juridiquement, constituent néanmoins un prix raisonnable pour obtenir un compromis avec l'Assemblée nationale sur l'adoption du texte. Je regrette toutefois que, dans une certaine mesure, la qualité de la loi soit la victime collatérale de l'accord que je vous propose. La parole est à M. Jean-Luc

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la proposition de loi examinée aujourd'hui en deuxième lecture nous redonne l'occasion d'évoquer le sujet essentiel de la lutte contre les décès consécutifs à un arrêt cardiaque et de la sensibilisation de nos concitoyens aux gestes qui sauvent. Cela a été rappelé, entre 40 000 et 50 000 personnes sont victimes, chaque année, d'un arrêt cardiaque, ce qui représente environ 120 décès par jour. Un tiers de ces victimes sont âgées de moins de 60 ans.

s'il est important de souligner que le délai d'action des secours est déjà très court- environ treize minutes, en moyenne -, l'enjeu est d'accroître sensiblement le nombre d'interventions de personnes ayant bénéficié de la formation aux premiers gestes qui sauvent et se trouvant à proximité immédiate de la victime. Cela nous permettrait de nous rapprocher des taux de survie de 20 % à 40 % observés dans les pays anglo-saxons et scandinaves, où les citoyens sont massivement formés au massage cardiaque. La formation aux gestes de premiers secours doit être fortement améliorée dans notre pays ; moins de la moitié des Français y est initiée, alors même qu'une formation de ce type est simple à suivre et peu onéreuse et qu'elle peut être reçue sur une période très brève. En quelques heures, il est effectivement possible de se familiariser avec la pratique d'un massage cardiaque, la mise en position latérale de sécurité ou le maniement du défibrillateur. Selon la Croix-Rouge, si l'on doublait le nombre de personnes formées au massage cardiaque, 2 000 vies pourraient être sauvées chaque année. Des initiatives innovantes, issues de la société civile, se sont d'ores et déjà développées, telles que des applications, comme « SAUV Life » ou « Permis de sauver

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a pris en considération une partie importante des apports et modifications sénatoriaux, tout en rétablissant plusieurs mesures, dont la portée symbolique paraissait importante, sans nuire à l'efficacité du texte. L'expression de « citoyen sauveteur » a notamment été maintenue, ce que je soutiens pleinement, ayant moi-même déposé deux amendements en ce sens en première lecture. En effet, que, tout en respectant l'encadrement juridique lié à cette nouvelle implication en tant que sauveteur, cette appellation permet de concourir à l'affirmation du sentiment d'appartenance à la communauté nationale.

la dimension citoyenne nécessaire pour réaliser cette ambition concrète de sensibiliser davantage la population aux gestes qui sauvent. Ont également été rétablies les dispositions relatives à l'instauration d'une journée nationale de lutte contre l'arrêt cardiaque, ainsi que la sensibilisation des élèves du second degré aux gestes qui sauvent. Je souscris pleinement à ce rétablissement ; j'avais, pour ma part, proposé de réintroduire un module d'apprentissage des gestes de premiers secours dans le cadre de la journée défense et citoyenneté. dit, nous nous rejoignons quant aux objectifs et je me félicite de l'instauration d'un continuum éducatif entre le premier degré et le second, qui favorisera un réel apprentissage des gestes de premiers secours. Par ailleurs, les salariés qui le souhaitent pourront également bénéficier d'une sensibilisation à ces gestes avant leur départ à la retraite, ce que je salue également. En effet, en la matière, nos concitoyens doivent pouvoir bénéficier d'une formation tout au long de la vie, avec des remises à niveau régulières, afin de ne pas perdre la maîtrise de ce qu'ils ont appris ; ils doivent également pouvoir bénéficier de l'apprentissage de nouvelles techniques. C'est d'ailleurs ainsi que le sentiment d'appartenance à la communauté des citoyens sauveteurs prendra tout son sens.

en faveur d'une meilleure formation de nos concitoyens à ces gestes essentiels, qui permettent de sauver des vies. La parole

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui en deuxième lecture prévoit de mieux former les Françaises et les Français aux réflexes de premiers secours, tout au long de leur vie, et de créer un statut de « citoyen sauveteur

le citoyen est le premier maillon de la chaîne des secours. » Selon les chiffres de la Fédération française de cardiologie, sans une prise en charge immédiate, plus de 92 % des arrêts cardiaques sont fatals. Dans sept cas sur dix, l'arrêt cardiaque survient devant des témoins, mais seulement 40 % de ceux-ci

D'après l'Association française des premiers répondants, l'AFPR, une question revient souvent lors des présentations au grand public des gestes de secourisme, celle des risques encourus si la victime vient à décéder ou présente des séquelles irréversibles malgré l'intervention d'un sauveteur occasionnel. Ainsi, la création du statut de « citoyen sauveteur », visant à protéger juridiquement les personnes qui pratiquent les premiers secours- en particulier le massage cardiaque -en modelant un régime de responsabilité favorable à l'intervention, représente une avancée importante. À cet égard, nous saluons le

Donner un véritable statut à ces citoyens responsables -je pense, comme Jean-Luc Fichet, que l'emploi du terme « citoyen » correspond tout à fait à l'esprit de cette loi -est donc bienvenu, mais il nous faut tout autant

La sensibilisation des élèves au secourisme et le droit à la formation aux premiers secours pour tout salarié sont, certes, déjà prévus par les règlements en vigueur, mais ils mériteraient d'être plus largement diffusés et mis en oeuvre. Nous avons des marges de progrès, tant l'apprentissage de ces gestes constitue aussi d'entrée dans la citoyenneté. Nous devons absolument mettre en place une politique ambitieuse et cohérente, permettant aux individus d'être formés lors de toutes les grandes étapes de la vie. Il s'agit d'un sujet tout à fait fondamental pour l'ensemble de nos concitoyens, notamment pour ceux

Plus encore, l'apprentissage de ces gestes a vocation à faire partie intégrante du bloc de compétences citoyennes à définir pour développer le sens de la citoyenneté et la cohésion sociale. Se savoir en capacité de sauver

déjà assez remarquable, mais il existe là aussi de véritables fractures territoriales : les temps d'intervention ne sont pas les mêmes en ville et

La proposition de loi, dans la rédaction que nous examinons aujourd'hui, résultant d'un compromis sur le fond entre nos deux chambres, favorise une faculté d'assistance réciproque, qui fait pleinement sens dans notre pacte social.

Je veux saluer l'accord dont ce régime équilibré, pierre angulaire du texte, a fait l'objet entre les deux assemblées. Une telle démarche a pour effet utile de garantir une meilleure accessibilité du droit pour les personnes mises en cause et d'assurer la sécurité juridique

Je remercie Mme la rapporteure d'y avoir consenti en deuxième lecture. Le texte vise ensuite à renforcer les dispositifs de sensibilisation aux gestes qui sauvent, construisant ainsi un vecteur de solidarité entre les citoyens. Cette sensibilisation n'est pas négligeable, puisque pas négligeable, puisque personne n'est à l'abri du risque d'arrêt cardiaque inopiné ; chaque citoyen constitue un maillon de la chaîne de survie et peut être appelé, en toutes circonstances, à se draper des habits du sauveteur, bien avant l'arrivée des secours.

continuum de formation aux gestes qui sauvent entre plusieurs lieux structurant la trajectoire de la majorité de nos concitoyens : l'école, le club sportif ou encore l'entreprise. Je vous sais réservée, madame la rapporteure, pour des raisons de droit que nous entendons bien, sur la création d'une journée nationale dédiée.

Les indicateurs mentionnés pourraient permettre d'identifier clairement les facteurs expliquant que, dans notre pays, l'arrêt cardiaque inopiné cause encore entre 40 000 et 50 000 décès par an. je veux souligner deux dispositions dont on ne peut nier la portée pratique : le renforcement des peines prévues en cas de vol ou de dégradation de défibrillateur et la faculté d'encadrement de la formation aux premiers secours,

À l'issue de son adoption conforme par la commission des lois, sur la proposition de la rapporteure, dans une version dont le Sénat a conforté l'assise juridique, cette proposition de loi est de nature à faire honneur au triptyque évoqué par son auteur : elle encourage, elle désacralise, elle protège mieux.

sauveteurs est donc indispensable si l'on veut réduire de manière significative le nombre des décès par arrêt cardiaque. En avril 2017, le rapport Faure-Pelloux s'inquiétait de ce que le taux de formation de la population française dans ce dans ce domaine soit parmi les plus faibles au monde. Il préconisait d'atteindre un taux de formation de la population de 80 %, et l'Académie nationale de médecine a confirmé cette préconisation dans son rapport du 2 octobre dernier. proposition de loi s'inspire directement de ces préconisations. Par conséquent, nous ne pouvons qu'en partager les objectifs, consensuels sur l'ensemble des travées : il s'agit de sensibiliser aux gestes qui sauvent et créer, conformément au souhait des professionnels de santé, un statut de

Derrière cette unanimité se cachent pourtant quelques questions. Il faut notamment souligner que, pour atteindre les objectifs ambitieux de formation fixés par le rapport Faure-Pelloux, il conviendrait d'impliquer de nombreux intervenants dans la chaîne de formation je pense en particulier aux enseignants et au personnel de santé, dont les tâches sont pourtant déjà bien lourdes. Sur le fond, si les premières minutes suivant un accident cardiovasculaire majeur sont décisives, nous ne perdons pour autant pas de vue que la survie du patient dépend aussi de la fiabilité de toute la chaîne d'intervention. Or celle-ci est particulièrement affaiblie. Les pompiers ont ainsi largement manifesté pour dénoncer un déficit de financement de l'ordre de 60 000 à 80 000 euros par caserne

du débat sur la crise de la Covid-19 semble déjà bien loin ; nos concitoyens et les soignants continuent de réclamer « du fric pour l'hôpital public Il faut bien l'avouer, la situation reste extrêmement tendue et ne permet pas de garantir une chaîne de soins qui soit digne d'un pays comme le nôtre. Nous prenons donc ce texte comme un premier pas,

Je peux d'autant mieux en témoigner que je suis moi-même engagé dans une démarche visant à atteindre cet objectif, au travers de l'utilisation de l'application « SAUV Life », lancée en 2018 et que j'ai connue ici, au Sénat, à une réunion organisée par une collègue sénatrice de la région parisienne, très mobilisée pour le développement et la promotion de cette application. Des dizaines de vies ont déjà été sauvées grâce à « SAUV Life » et plusieurs milliers de personnes font aujourd'hui partie de cette communauté. Grâce à cette application, des sauveteurs amateurs, géolocalisés dans un périmètre restreint, sont alertés leur téléphone portable pour venir en aide à une personne en situation d'arrêt cardiaque. Figurez-vous qu'il m'est arrivé d'être sollicité alors même que je participais à une réunion dans la salle Monory, j'ai été alerté pour venir en aide à une personne résidant dans un immeuble de la rue Madame, à 500 mètres du Sénat. Je suis arrivé sur place en même temps que les pompiers, mais avant

relatifs à l'obligation de formation au secourisme, sont intéressants. Le premier de ces articles concerne spécifiquement les juges et arbitres de fédération sportive et le second a trait à la formation par certains acteurs de santé. Chaque Français doit avoir conscience qu'il est un acteur potentiel de la solidarité nationale

également rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, est à la fois clair et louable. Il s'agit d'attirer l'attention sur le sujet majeur de l'arrêt cardiaque,

Il est à noter que le dispositif dont nous sommes amenés à discuter aujourd'hui trouve déjà à s'appliquer dans de nombreux pays étrangers : aux États-Unis, dans plusieurs provinces du Canada, en Australie, en Finlande ou encore en Allemagne. La loi communément appelée « », ou « loi du bon Samaritain », comporte un ensemble de dispositions destinées à protéger les citoyens, en particulier les secouristes bénévoles qui portent assistance, contre d'éventuelles poursuites judiciaires. Par exemple, l'article 1471 du code civil du Québec précise que la personne qui porte secours à autrui est exonérée de toute responsabilité pour le préjudice qui peut en résulter, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa

plus juridique, de « sauveteur occasionnel et bénévole », qui nous paraissait davantage appropriée s'agissant d'un concours apporté à l'exercice d'un service public. Cependant, le rapporteur de l'Assemblée nationale a clarifié la manière dont cette expression devait être entendue : ce statut recouvre l'acte de civisme commis par un citoyen qui porte

au secourisme pour les juges et arbitres des fédérations agréées ou à l'introduction dans le code pénal de circonstances aggravantes relatives au vol ou à la destruction, détérioration ou dégradation de matériels destinés à prodiguer

Enfin, d'autres réintroductions d'articles, qui, au départ, ne nous semblaient pas souhaitables sur le fond, nous paraissent aujourd'hui permettre un compromis acceptable entre les deux chambres du Parlement sur cette proposition de loi. Je reviendrai notamment sur l'article 6, tendant à créer une journée nationale de lutte contre l'arrêt cardiaque et de sensibilisation aux gestes qui sauvent.

un consensus intelligent, en élaborant un texte qui dépasse les clivages politiques. Je salue la volonté de tous les élus de se saisir du sujet de santé publique majeur qu'est l'arrêt cardiaque inopiné et de sensibiliser le plus grand nombre de nos concitoyens

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, selon la Fédération française de cardiologie, sans prise en charge immédiate, plus de 90 % des arrêts cardiaques sont fatals. Leur prise en charge a été systématisée par une chaîne de survie. Après un arrêt cardiaque, chaque minute compte et la réalisation de gestes le plus tôt possible permet d'augmenter au maximum les chances de survie de la victime. La première étape consiste à appeler les secours ; la deuxième, à pratiquer un massage cardiaque ; la troisième, à faire usage d'un défibrillateur ; la quatrième, à prodiguer des soins spécialisés à la victime jusqu'à la reprise de respiration ou à l'arrivée des secours. La proposition de loi qui est soumise à notre examen aujourd'hui a été adoptée en deuxième lecture par l'Assemblée nationale. Elle s'organise autour de trois axes : créer un statut de citoyen sauveteur, pour identifier et protéger celui qui porte secours aux victimes mieux sensibiliser la population aux gestes qui sauvent ; clarifier l'organisation des différentes sensibilisations et formations aux premiers secours. Sept fois sur dix, les arrêts cardiaques surviennent devant témoins, mais seulement 40 % de ceux-ci accomplissent les gestes de premiers secours. La conséquence en est que, en France, le taux de survie à un arrêt cardiaque ne dépasse pas les 8 %, alors qu'il est de quatre à cinq fois plus élevé dans les pays où les lieux publics sont équipés en défibrillateurs automatisés externes et où la population est formée aux gestes qui sauvent. Chaque minute qui passe avant l'arrivée des secours, c'est 10 % de chances de survie en moins. Les premiers secours, c'est à la fois une formation, des acteurs, du matériel et des modalités.

Comme le précise le docteur Lionel Lamhaut, médecin au SAMU de Paris et cofondateur de l'application, ce sont près de 350 000 citoyens sauveteurs répartis sur l'ensemble du territoire qui sont inscrits sur cette application et plus de quatre-vingt-cinq coeurs qui ont ainsi pu repartir. Je souhaite ajouter quelques mots à propos de la crise de la Covid-19. Afin d'éviter un effondrement du système de santé pendant le pic de l'épidémie, le Plan blanc a été déclenché sur l'intégralité du territoire, ce qui a notamment conduit à l'annulation de soins et d'interventions programmés et au report de consultations jugées non essentielles. De nombreux Français souffrant de maladies chroniques, dont des pathologies cardiaques structurelles, ont ainsi reporté des soins pourtant nécessaires hésitent encore à se rendre chez leur médecin ou à l'hôpital. Or, au regard de la Covid-19, ces personnes concentrent les facteurs de risque, en raison de leur âge et de l'impact du virus sur l'appareil cardiovasculaire.

est suspendue. La séance est reprise. J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la délégation sénatoriale aux entreprises a été publiée. Cette candidature sera ratifiée si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement.

Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses, dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Je rappelle que l'auteur de la demande dispose d'un temps de parole de huit minutes, puis le Gouvernement répond, pour une durée équivalente. À l'issue du débat, l'auteur de la demande dispose d'un droit

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui pour débattre d'un sujet majeur et plus que jamais d'actualité. La délégation aux entreprises du Sénat s'en est saisie à l'automne 2019, en confiant à nos collègues Michel Canevet et Guy-Dominique Kennel une mission d'information sur les difficultés de recrutement dans un contexte de forte évolution des métiers.

à trouver et à garder les compétences dont ils avaient besoin, cette situation les amenant parfois à renoncer à développer leur activité. Parallèlement, la France pouvait rougir de son taux de chômage et du nombre de personnes, notamment des jeunes, laissées au bord de la route. Quel gâchis ! route. Quel gâchis ! Les mutations technologiques qui impactent ou impacteront quasiment tous les métiers renforcent l'urgence de prendre à bras-le-corps ce paradoxe français, avec lucidité et bon sens. L'électrochoc que nous connaissons aujourd'hui a le mérite de nous encourager, collectivement et individuellement, à remettre les cartes sur la table, à évaluer nos atouts et nos faiblesses, à retrousser nos manches, à oser, à innover et à jouer franc-jeu avec toutes les parties prenantes. le cas présent, ces dernières comprennent les acteurs de l'éducation, de l'orientation des jeunes et du service public de l'emploi, les régions, les demandeurs d'emploi, les personnes en future reconversion et, bien entendu, les recruteurs eux-mêmes, c'est-à-dire les entreprises au premier chef. À cet égard, l'État doit aussi aider les entreprises à contribuer à la formation de leurs salariés ou futurs salariés. Un très récent sondage réalisé pour montre que 13 % des entreprises n'envisagent pas de mettre en place de contrats d'alternance dans l'année à venir, car les modalités de prise en charge financière sont trop compliquées. Je crois pouvoir dire que, au sein de notre délégation, nous partageons la conviction que la clé de l'avenir passe par le renforcement des compétences des Français. Il s'agit à la fois de permettre leur insertion et leur épanouissement professionnels tout au long de la vie et de répondre aux besoins de la société et de l'économie, les deux étant bien sûr liés. Nos propositions visent ainsi à développer les compétences de toute urgence pour soutenir l'emploi et les entreprises. Certes, depuis l'automne 2019, la situation sanitaire et économique a bouleversé la donne. Les chiffres ne sont pas réjouissants : probable recul de près de 12 % du PIB en 2020, déficit budgétaire de 221,1 milliards d'euros, dette publique s'élevant à 120,9 % du PIB, nombreuses faillites en perspective L'horizon s'assombrit, avec la perspective de la suppression de 800 000 emplois, soit 2,8 % de l'emploi total, dans les prochains mois. Mais la problématique des jours d'avant le Covid-19 reste cruellement d'actualité. Elle se conjugue avec les nouveaux défis des jours d'avec et des jours d'après la crise sanitaire, qu'accompagne et suit la crise économique. Il est vrai que les dispositifs de soutien très évolutifs mis en place depuis le début de la crise devraient permettre de limiter et de lisser la casse économique et sociale,

à la fois pour limiter la casse sociale et pour préparer l'avenir. Cette crise doit être l'occasion de remettre en cause certains tabous et d'avancer collectivement dans l'intérêt général et dans celui des personnes concernées

Trois nécessités se sont dégagées à l'issue de nos travaux : accompagner les individus tout au long de la vie et lors de la formation initiale, avec pour objectif constant d'améliorer leur insertion professionnelle et leur employabilité employabilité ; permettre aux entreprises de trouver rapidement les compétences dont elles ont besoin ; définir les modalités d'un pilotage efficient des acteurs de l'emploi sur chaque territoire.

accentuer les efforts d'information des familles en vue de l'orientation des jeunes et permettre aux enseignants de mieux appréhender les questions économiques et la vie des entreprises.

Ces travaux, qui ont débuté en septembre dernier, nous donnent l'occasion aujourd'hui d'alimenter les réflexions en cours, notamment avec les partenaires sociaux, sur un sujet essentiel qui nous mobilise toutes et tous, à savoir l'emploi et les compétences. Lorsque la situation était meilleure, cette mobilisation était nécessaire pour trouver les compétences que recherchaient les entreprises. Elle est aujourd'hui un élément clé de la relance. Le sujet des emplois et des compétences est ma priorité.

et celle d'un véritable conseil en évolution professionnelle. Nous avons amplifié massivement l'accès à la formation grâce à l'application « Mon compte formation », qui connaît un succès très important et croissant.

À cet égard, il convient de souligner que notre action pour soutenir les entreprises et les salariés les plus précaires pendant les périodes de confinement et de déconfinement a été déterminante.

L'État a, de fait, pris en charge automatiquement 100 % des coûts pédagogiques, sans plafond horaire, compte tenu de la crise. Nous constatons une dynamique intéressante : plus de 120 000 salariés sont désormais en formation grâce à ce dispositif. Parallèlement, plus de 50 000 personnes ont formulé

Enfin, le télétravail a permis à des millions de Français de poursuivre leur activité, mais aussi de se former. Je rappelle que c'est un droit pour le salarié, que nous avons créé en 2017, au travers des ordonnances « travail ». Plus que jamais, dans la nouvelle phase, celle de la reprise de l'activité, nous partageons ce constat : nous devons tout faire pour préserver nos emplois et nos compétences. est notre priorité commune, à l'heure où les circonstances nous appellent à reconstruire une économie forte, écologique, souveraine et solidaire, comme l'a déclaré le Président de la République dans sa dernière allocution.

S'agissant de la recommandation n° 13, sur la nécessité de sensibiliser les PME à l'absence de candidat idéal et aux atouts de la formation professionnelle, sa mise en oeuvre se concrétise à travers différents moyens

à notre demande, le règlement de l'Autorité des normes comptables permet dorénavant aux entreprises de pratiquer, sur option, l'amortissement des frais de formation liés à l'acquisition d'une immobilisation corporelle ou incorporelle.

Nous partageons également votre souhait d'une meilleure rentabilisation de la data en matière d'emploi ; vos trois recommandations en ce sens sont très importantes. Par ailleurs, je rappelle que, dès cet été, l'intégration de Pôle emploi au dispositif « Mon compte formation » permettra des abonnements complémentaires.

au débat interactif. Je rappelle que chaque orateur dispose de deux minutes au maximum pour présenter sa question, avec une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente. Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires, à la condition que le temps initial de deux minutes n'ait pas été dépassé.

je voudrais souligner une difficulté émergente, qui, selon moi, va s'accentuer fortement : le refus croissant des jeunes diplômés de travailler pour des entreprises ne correspondant pas à leurs valeurs en termes environnementaux et sociaux. Voilà un an, des jeunes issus de grandes écoles, réunis au sein du collectif « Pour un réveil écologique », ont lancé un manifeste, signé par plus de 32 000 étudiants de grandes écoles écoles s'engageant à refuser de rejoindre des entreprises polluantes. Cette initiative est révélatrice d'une tendance de fond : selon une étude de la Confédération des grandes écoles, 72 % des jeunes considèrent l'adéquation entre travail et

il est pertinent d'adapter les compétences de la population aux entreprises, mais ne doit-on pas également inverser la logique, ou plutôt rétablir l'ordre des choses ?

et à amorcer des politiques de formation anticipant les transitions de nos sociétés. C'est ainsi que nous ferons face aux menaces liées au réchauffement climatique et à l'effondrement de la biodiversité ! La parole

ils ne veulent pas d'un bureau classique et indiquent souvent qu'ils choisiront une entreprise qui leur permettra de télétravailler. Cette génération demande une meilleure prise en considération de ses conditions de travail, en particulier un équilibre plus juste entre vie professionnelle et vie personnelle.

consacrant chaque jour environ une heure à ces trajets ; sur une année, ce sont plus de 6 milliards d'heures de déplacement. Pendant la crise sanitaire que nous venons de vivre, le recours au télétravail a été massif.

En réalité, cette crise sanitaire va très certainement changer nos rapports au travail et à l'entreprise : en bref, plus de télétravail et des Français plus désireux d'y recourir.

d'information. De ce point de vue, le sort réservé aux lycées et à l'enseignement professionnels est inquiétant : moins d'heures d'enseignement général, moins d'enseignements professionnels, des programmes tirés vers le bas, autant d'éléments

du monde de l'entreprise ... La réforme de l'apprentissage que vous avez engagée, madame la ministre, renforce ces craintes. En effet, confier cette voie aux seules branches professionnelles laisse place à une vision court-termiste

de ces formations. D'ores et déjà, des entreprises alertent à cet égard. Nous avons besoin de tout l'engagement de la puissance publique, d'un État stratège capable d'identifier les secteurs d'avenir et de développer les formations adéquates.

Les réformes commençaient à porter leurs fruits, et l'objectif d'un taux de chômage ramené à 7 % à la fin du quinquennat paraissait, voilà quelques mois encore, réaliste. Nous aurions tort de baisser les bras : la France ne doit jamais se résigner au chômage de masse, souvent perçu comme une fatalité nationale.

La lutte contre le chômage doit devenir « verte », et l'écologie devenir la solution aux problèmes de recrutement des entreprises ! Il s'agit de mettre fin à ce paradoxe aberrant, malheureusement propre à la France : des demandeurs d'emploi ne trouvent pas de travail et des entreprises ne trouvent pas d'employés ... Une relance verte implique une évolution importante du marché de l'emploi. En effet, les entreprises devront décarboner leur modèle économique, nous devrons amplifier la rénovation énergétique du parc immobilier, nos mobilités seront progressivement bouleversées et nous aurons besoin de développer de nouvelles compétences, adaptées à de nouveaux métiers. Tout cela est évident,

compte-t-il articuler lutte contre le chômage et lutte contre le changement climatique ? Quel est son plan d'action pour mener ces deux combats de front, étant entendu que nous ne pouvons renoncer ni à l'un ni à l'autre ? La parole est à Mme la ministre. Monsieur le

ont concouru à faciliter la reconversion. Grâce à leurs compétences économiques et à leur connaissance du tissu entrepreneurial, les régions ont pu agir positivement. Pourtant, les dernières tentatives de décentralisation se sont montrées inefficaces, parce qu'elles n'ont été que partielles. Ainsi, la non-concrétisation du transfert de Pôle emploi vers les régions du pilotage de l'achat des formations pour demandeurs d'emploi empêche aujourd'hui d'envisager toutes les formations à l'aune des besoins en compétences locaux. Combien de temps encore maintiendra-t-on cette multiplicité des commandes de formations à destination des demandeurs d'emploi, émanant de Pôle emploi, des OPCO, des régions, de

L'urgent défi serait plutôt d'en juguler les conséquences sociales, donc de renoncer d'abord aux ordonnances inhumaines sur le chômage. Pour autant, l'adéquation entre offre et demande d'emploi reste une question récurrente, de vue des statistiques, qui ne varieraient pas beaucoup, que de celui du dynamisme des entreprises. Citons quelques obstacles semés sur la route des recruteurs : une trop grande exigence de technicité par rapport au vivier des candidatures,

La mission El Khomri montre un déficit en candidatures de personnels de santé lié aux rémunérations trop basses. Les difficultés d'accès au lieu de travail et les temps partiels ou saisonniers sont également très dissuasifs. Notons également que, depuis 2015, l'offre de CDI augmente régulièrement et allonge le temps de recrutement. En conséquence, madame la ministre, un certain nombre de pistes peuvent être dégagées : inciter à une meilleure formation théorique et intellectuelle pour plus d'adaptabilité éviter les offres de CDD trop courts, donc développer les temps complets par des groupements d'employeurs et la création- pourquoi pas ? -d'agences publiques, pour multiplier les CDI d'intérim ; encourager dans les négociations de branche une attitude bienveillante et accompagnante dans les entreprises pour une adaptation au poste de travail ; enfin, mobiliser des dynamiques de bassin entre villes et campagnes pour créer les outils de prévision des besoins à venir, tant du privé ou du public que des associations, et ainsi engager les formations utiles. Les spécificités locales, particulièrement marquées dans le domaine de l'économie, donc de l'emploi, exigent une nouvelle phase de décentralisation, une véritable décentralisation pour une nouvelle vitalité des territoires.

M. Michel Canevet. Si la question de l'acquisition des compétences par la formation, qu'elle soit initiale ou continue, est absolument cruciale pour apporter une réponse aux besoins évolutifs de l'entreprise de demain,

je félicite Michel Canevet et Guy-Dominique Kennel de la qualité de leur rapport et je les remercie d'avoir abordé la question de la numérisation de notre économie et des difficultés de recrutement qui en découlent. Notre pays accuse un retard dans ce domaine. Avec 191 000 postes à pourvoir d'ici à 2022, la France connaît une réelle pénurie de compétences en matière numérique. Plus grave encore : l'illectronisme touche près de 20 % de nos concitoyens. Ce constat appelle des mesures fortes. La première urgence est de renforcer l'information du grand public en inscrivant le numérique dans la logique du système éducatif, sur le modèle des pays nordiques. L'apprentissage des usages du numérique doit aller de pair avec celui de la lecture. D'autres pistes doivent être explorées, comme la systématisation de l'évaluation numérique de tous les enseignants et élèves, ou encore la création d'un baccalauréat professionnel « services numériques On retrouve bien sûr ce manque de compétences numériques au sein de l'entreprise. Beaucoup de dirigeants de PME n'ont pas conscience de la nécessité de se former eux-mêmes ou de former leurs salariés, d'où l'importance d'insuffler une vraie culture de formation numérique des salariés pour garantir leur employabilité. L'incitation financière pourrait à ce titre constituer un premier socle pour changer les comportements, par exemple par la création d'un suramortissement des investissements réalisés en vue d'améliorer les compétences, compétences, d'un crédit d'impôt spécifique ou d'une réduction du montant de la taxe d'apprentissage pour les entreprises qui font l'effort de former leurs salariés. La reconversion numérique des chômeurs est aussi un moyen de pallier la pénurie de main-d'oeuvre. Le numérique et internet rassemblent en effet le premier contingent d'offres de recrutement, devant la santé et l'action sociale. Ma question est donc simple : quelles initiatives le Gouvernement entend-il prendre pour diffuser partout et pour tous une véritable culture du numérique, et ainsi faire entrer la France dans la quatrième révolution industrielle ? La parole est à Mme la ministre.

donc l'appropriation par tous du numérique. Quelles sont les actions que menons ? Tout d'abord, dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences et de la grande école du numérique financée par l'État, nous avons lancé un grand appel à projets pour mettre en place 10 000 formations numériques à tous niveaux.

le Président de la République a récemment plaidé pour la reconquête de la souveraineté économique de la France et la relocalisation d'activités stratégiques sur le territoire national. Cette volonté politique s'inscrit dans le cadre d'une réflexion plus large sur la réindustrialisation de notre pays et la relocalisation des emplois.

n'est-ce pas une gageure que de vouloir réindustrialiser à tout prix, avec la fausse bonne idée que cette politique permettra de traiter la question du chômage, notamment celui des jeunes, et celle du retour à la prospérité économique ? Ce serait méconnaître que, à 80 %, la perte d'emplois industriels est liée au progrès technique, et que les délocalisations ont répondu à une logique économique. Ce serait également méconnaître que le faible poids de l'industrie dans notre pays est la conséquence du manque de compétences industrielles. Nos entreprises peinent à se développer parce qu'elles ne trouvent pas les compétences et les capacités dont elles ont besoin dans un certain nombre de spécialités. Nous formons par exemple deux fois et demie moins d'ingénieurs en France qu'en Allemagne. L'industrie de demain sera celle des robots d'intelligence artificielle. La question de la formation est donc majeure. Florent Menegaux, président de Michelin, a rappelé récemment que nous formons nos élites à des technologies et à un environnement économique du passé, et qu'un travail très important doit être réalisé dans ce domaine. Madame la ministre, je vous poserai donc trois questions. Tout d'abord, aussi louable que soit l'ambition de réindustrialiser notre pays, comment comptez-vous procéder pour adapter le système éducatif, aujourd'hui à la peine, au besoin des entreprises industrielles de demain ? Ensuite, envisagez-vous d'encourager puissamment les formations scientifiques et d'ingénieur, susceptibles d'offrir à ces entreprises les profils et les compétences recherchées ? Enfin, comment favoriser une plus grande interaction avec le monde de l'entreprise, où, comme le dit fort justement le président de Michelin, l'on doit marier la théorie à l'expérience en la confrontant à la pratique ? La parole

plus limité. Tous les grands groupes industriels, ou quasiment, sont en train de développer l'apprentissage, ce qu'ils n'arrivaient pas à faire auparavant, parce qu'ils veulent créer les compétences de demain. Contrairement à ce que disait M. Tourenne,

Par ailleurs, on assiste à une prise de conscience généralisée, en particulier de la jeunesse, sur la nécessité d'une transition écologique pour réduire l'impact de l'activité humaine sur notre environnement. N'en doutons pas, ces deux transitions sont en cours et auront des répercussions, tant sur les métiers que sur les formations. Je partage dès lors l'analyse de nos collègues rapporteurs, selon laquelle le recrutement, notamment des jeunes, doit être au coeur de nos préoccupations. Le contexte actuel rend d'autant plus insupportable le constat, qui est dressé dans ce rapport, de difficultés de recrutement liées à une inadéquation entre le profil des candidats et le poste. Qui mieux que les acteurs locaux peut pallier une telle difficulté ?

De la même manière, il me semble opportun d'encourager la coconstruction par les établissements d'enseignement supérieur, dont on parle peu, et les acteurs locaux d'une offre de formation qui corresponde exactement aux besoins spécifiques du territoire. À ce titre, les campus des métiers et des qualifications sont des dispositifs qui méritent, me semble-t-il, d'être renforcés. Ce label permet d'identifier, sur un territoire donné, tout un réseau d'acteurs qui interviennent en partenariat pour développer une large gamme de formations professionnelles, technologiques et générales, centrées sur des filières spécifiques et sur un secteur d'activité correspondant à un enjeu économique régional. Dans un contexte où tant l'enseignement supérieur que le marché du travail vont connaître d'importantes mutations, mettre tous ces acteurs autour de la table me semble pertinent.

on l'a vu récemment lors de la crise sanitaire, il y a aussi des jeunes qui se sont investis et dévoués. On sait que la tâche

Mme la ministre.

qui, à part, les dirigeants et les salariés, le sait ? Les entreprises de ce département ont besoin de main-d'oeuvre pour exercer tous les métiers, du plus simple au plus spécialisé. Pourtant, même les enfants de nos territoires ignorent ce qu'il s'y passe vraiment. En même temps, je les pardonne : ils n'y sont pour rien ; c'est simplement parce que leur cursus scolaire ne le permet pas. Je pense que l'orientation est la solution à condition qu'elle se fasse en partenariat avec les entreprises. Dès la troisième, les collégiens devraient découvrir les métiers qui leur sont offerts sur leur territoire, et à plusieurs reprises. L'éducation nationale ne doit dorénavant plus ignorer la vie économique d'un territoire, et le monde économique doit aussi saisir cette chance. C'était le premier point Par ailleurs, je suis chef d'entreprise. Comme mes collègues, nous avons négligé l'accueil des jeunes et la formation à cause des contraintes imposées par l'inspection du travail à une époque, il faut le rappeler. Mais nous sommes conscients qu'une entreprise n'a pas d'avenir si elle ne forme pas. L'alternance et l'apprentissage à tous les niveaux sont donc d'excellentes choses que nous devons encourager. Pour accélérer ce processus, ne serait-il pas opportun d'appliquer une réduction sur la taxe sur les salaires pour ceux qui forment et qui forment bien, et, inversement, d'appliquer une majoration pour ceux qui ne forment pas

Ce n'était pas dans votre question, mais j'ai envie de le dire à cette occasion : avec ce que l'on vient de vivre depuis trois mois, je pense qu'il va se passer des choses en matière d'aménagement du territoire, non pas parce que nous le décidons, mais parce qu'un certain nombre de gens ont décidé qu'ils veulent vivre autrement.

J'ai compris qu'elles avaient été lues : j'espère qu'elles seront pour certaines entendues, voire traduites dans les faits. Je voudrais vous donner deux ou trois exemples. Tout d'abord, la délégation est exemplaire, parce qu'elle intègre elle-même un apprenti

je dois vous dire que je suis heureux que l'on découvre enfin les vertus de l'apprentissage. J'ajoute que les propositions qui ont été faites ici, dans cet hémicycle, la loi sur l'apprentissage de 2016, étaient vraiment concrètes ; certaines ont été reprises par le Gouvernement, ce dont nous nous réjouissons. Comme quoi, le Sénat peut offrir des propositions intéressantes. Madame la ministre, vous avez qu'un certain nombre d'outils existent déjà. Je vais parler de l'orientation : j'en suis désolé, mais l'orientation n'existe pas en tant que telle : les 54 heures

le souci de la réussite, celle des entreprises, évidemment, celle de nos territoires, mais aussi la réussite de l'ensemble de notre jeunesse. Et si nous proposons, par exemple, que la région